mes chers collègues, les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » demandés pour 2024 s’élèvent à 30,7 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. Les crédits de la mission augmentent de 4,6 % par rapport à la loi de finances pour 2023, poursuivant ainsi leur dynamique. La mission a en effet été fortement mobilisée ces dernières années. Il est ainsi permis de douter de la trajectoire définie dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 : les crédits de la mission ne devraient en effet augmenter que de 5 % en termes réels à l’horizon 2027. Compte tenu des exercices passés, il est probable que le respect de cette trajectoire dépende d’aléas conjoncturels. Je souhaite dire un mot de l’aide alimentaire, qui ne représente, avec 142 millions d’euros, qu’une faible part des crédits de la mission, mais qui constitue une politique vitale pour nombre de nos concitoyens, particulièrement en période inflationniste. Cette année, la situation des associations d’aide alimentaire est particulièrement inquiétante. Plus de 200 000 nouveaux bénéficiaires ont été accueillis, alors que l’inflation continue de peser sur les capacités des associations : le budget d’achat de denrées des Restos du Cœur, par exemple, a doublé en un an L’augmentation des crédits d’aide alimentaire dans le présent projet de loi de finances, qui concerne principalement le plan « Mieux manger pour tous », ne constitue pas une réponse adaptée à l’urgence. Heureusement, le Parlement a ouvert 40 millions d’euros supplémentaires dans la loi de finances de fin de gestion pour 2023 – 20 millions sur l’initiative de l’Assemblée nationale et 20 millions sur celle du Sénat – pour combler les lacunes du Gouvernement. Ce budget témoigne également d’un renouvellement du partenariat entre l’État et les collectivités, en particulier les départements, dans le champ des politiques sociales. Le pacte des solidarités, qui prend la suite, à compter de 2024, de la stratégie nationale de comporte un volet contractualisé avec les collectivités, au travers des pactes locaux des solidarités. Pour 2024, 190 millions d’euros sont budgétés à ce titre dans la présente mission, 53 % de ces crédits étant destinés à la contractualisation, au premier chef avec les départements. Je suis satisfait de constater que certaines des recommandations que nous avions formulées l’année dernière, lors de notre contrôle de cette contractualisation, ont été suivies. Ainsi, davantage de place sera laissée aux initiatives locales et un financement pluriannuel est prévu pour améliorer la visibilité pour les départements. Je souhaiterais mentionner en conclusion deux points aveugles de ce budget. Le premier concerne la protection juridique des majeurs. Dans notre pays, le nombre de mesures de protection par mandataire est particulièrement élevé : on dénombre aujourd’hui en moyenne soixante mesures par mandataire, alors qu’il faudrait en compter environ quarante cinq pour un travail Le Gouvernement avait promis une augmentation de 200 ETP du personnel des services mandataires, mais les crédits ouverts à ce titre sont insuffisants. Des mesures devront être prises Le second concerne le soutien de l’État aux départements au titre de la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA). Les crédits alloués à ce titre diminuent, passant de 89 millions d’euros en 2023 à 67 millions d’euros Heureusement, le Gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités et de ramener le soutien de l’État à son niveau de 2023, au travers de l’amendement n° II 1027, auquel la commission se montrera favorable. Compte tenu des sommes en jeu, la commission propose d’adopter les crédits de cette mission.

Je pense notamment à la mise en œuvre, au 1 octobre 2023, de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Nous l’appelions de nos vœux depuis plusieurs années. Désormais, les revenus pris en compte pour le calcul de l’AAH ne comprendront plus ceux du conjoint ; c’est une très bonne chose. Ce sont ainsi plus de 40 000 bénéficiaires de l’AAH qui verront leur allocation augmenter, pour un montant moyen de 320 euros, et 80 000 personnes exclues du bénéfice de cette allocation qui pourront désormais la percevoir, pour un montant moyen de 370 euros. Aucun allocataire ne verra son AAH diminuer, grâce à une mesure de maintien du mode de calcul le plus favorable. Au total, le coût de la mesure serait de 83 millions d’euros en 2023 et de 500 millions d’euros en année pleine. En outre,

à bénéficier de leur allocation, lorsqu’ils décident de travailler après 62 ans. On leur donne ainsi le même choix qu’au reste de la population quant au moment opportun de prendre leur retraite. L’article 65 permet quant à lui aux bénéficiaires de l’AAH qui perdent le droit à cette allocation du fait d’une revalorisation de leur pension de continuer à percevoir la majoration pour la vie autonome ou le complément de ressources. La commission y est favorable.

d’une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales. La création de cette aide, inspirée d’expérimentations locales, notamment dans mon département du Nord, est très positive elle doit permettre d’apporter une réponse aux femmes qui ne peuvent quitter leur conjoint violent faute de moyens financiers suffisants. Le montant prévu à ce titre pour 2024 paraît un peu faible : seulement 13 millions d’euros. Il risque de n’être pas suffisant pour financer une aide de 607 euros par femme éligible. Le Gouvernement semble tabler sur un important non recours ou sur un faible montant pour cette aide universelle d’urgence. Toutefois, l’aide pourrait être modulée selon la situation des bénéficiaires. Surtout, elle pourrait prendre la forme d’un prêt remboursable par le conjoint violent, une fois celui ci définitivement condamné. Si cette modalité de financement prédomine, l’aide universelle d’urgence pourrait bien être fort utile, même si elle est dotée de moyens modérés. À ce titre,

s’élèvent à 30,85 milliards d’euros, en hausse de 4,64 % par rapport à 2023, sous l’effet notamment de la revalorisation des prestations sociales consécutive à l’inflation et de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés. Le budget de la mission pour 2024 permet au Gouvernement d’ouvrir plusieurs chantiers en matière de lutte contre la pauvreté, d’accompagnement par le travail des personnes en situation de handicap, ainsi que de lutte contre les violences conjugales. L’importance de ces enjeux doit nous conduire à suivre ces chantiers avec attention et exigence. Je pense d’abord à l’aide alimentaire, dont les crédits augmenteront de plus de 20 % en 2024. sociales a estimé que cela restait encore insuffisant pour répondre à l’augmentation des files actives et à l’apparition de nouveaux publics, puisque 10,7 % des personnes ayant recours à l’aide alimentaire ont un CDI.

Elle constate cependant avec satisfaction que ce pacte poursuivra la pratique de contractualisation avec les collectivités territoriales, à laquelle 53 % de ses crédits seront destinés. La commission se félicite également de la création, sur l’initiative du Sénat, d’une allocation universelle d’urgence pour les victimes de S’agissant des mineurs non accompagnés, la contribution de l’État aux dépenses des départements diminue de 22 millions d’euros, traduisant la baisse attendue des flux concernés en 2024.

au titre de la protection juridique des majeurs sont en hausse de 3,87 % ; ils doivent permettre de répondre à l’augmentation du nombre de mesures de tutelle et de curatelle due au vieillissement de notre population.

les crédits consacrés aux communications institutionnelles en faveur de l’égalité femmes hommes à leur niveau de 2023. Il aurait paru incompréhensible que, l’année où la France accueille les jeux Olympiques, cette enveloppe diminue de moitié, alors même que les risques accrus

de la mission. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps de l’intervention générale et celui de l’explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

s’intensifie et se féminise. Les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », en plus d’être notoirement insuffisants, prennent trop peu en compte les besoins financiers de la lutte contre contre la pauvreté, notamment celle des enfants, ainsi que de la réduction des inégalités entre femmes et hommes. Le constat de l’intensification de la pauvreté et de son élargissement est alarmant. Selon l’Insee, en France, au début de 2022, la proportion de personnes en privation sociale et matérielle a atteint son plus haut niveau depuis 2013 ; cette

Une personne sur quatre ne pouvait se payer une semaine de vacances dans l’année. Une partie de la population, plus importante d’année en année, n’a pas les moyens de s’acheter des vêtements neufs, de posséder deux paires de chaussures

ministres ! Dans le même temps, l’Unicef France publie un rapport sur l’état des droits des enfants dans les outre mer, où il est indiqué que « la pauvreté endémique [y est] responsable de conséquences multidimensionnelles ». Or, tandis que tous les besoins augmentent, les crédits ne suivent pas. Après une nette hausse du budget consacré à la protection de l’enfance, que nous avions saluée, nous regrettons que cette ligne connaisse cette fois une baisse de 5 %. Le PLF 2024 acte également la fin de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, remplacée

contre la pauvreté ». Plutôt que de proposer des mesures structurelles afin de réduire durablement la pauvreté, telle l’augmentation des minima sociaux, le pacte des solidarités propose un axe de « sortie de la pauvreté par l’activité et l’emploi », unique focale qui, dans un marché du travail dérégulé, fabriquera en grand nombre des travailleurs beaucoup le resteront durablement. Face à cette pauvreté, l’augmentation des crédits consacrés à l’aide alimentaire ne suit ni l’explosion des besoins ni l’inflation alimentaire dopée aux surmarges des grands groupes – un effet de ciseaux qui asphyxie les associations d’aide alimentaire. En France, un tiers de la population n’est pas en mesure de se procurer une alimentation saine en quantité suffisante pour trois repas par jour ; les banques alimentaires accueillent 34 % de

L’avis de la commission des affaires sociales le souligne : « à périmètre égal, c’est à dire sans la création de l’aide aux victimes de violences conjugales, les crédits seraient en baisse de 3,65

mes chers collègues, la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » finance l’ensemble des politiques en faveur des travailleurs pauvres, des enfants, des familles vulnérables, des personnes dépendantes ou en situation de handicap, de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le PLF 2024 prévoit une progression des crédits de la mission, de 1,3 milliard d’euros, mais cette hausse de 4,6 % doit être relativisée au vu du niveau de l’inflation, qui devrait atteindre 2,6 % l’an prochain. De fait, en euros constants, les crédits progressent seulement de 0,9 % en 2024, alors que 11 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté et que 2 830 enfants dorment dans la rue en France,

née de la pandémie, le Gouvernement a été capable de débloquer 200 milliards d’euros pour les entreprises. Aujourd’hui, alors que des millions de familles peuvent basculer dans la précarité, voire la grande précarité, seulement 1,3 milliard d’euros supplémentaires seront versés aux personnes handicapées, aux jeunes sans emploi et aux personnes vulnérables. Alors que toutes les associations signalent qu’elles sont confrontées à une augmentation sans précédent de demandeurs, seulement 142 millions d’euros sont prévus pour l’aide alimentaire. Les crédits de l’action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables », qui se montent

Cette année, les crédits de la mission traduisent également la création de l’aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales. C’est une bonne chose, mais, là encore, regardons avec attention cette avancée

! Plus globalement, le budget de la lutte contre les violences faites aux femmes, présentée comme une « grande cause » du quinquennat Macron, est largement insuffisant. En cinq ans, le budget affecté à la lutte contre les violences a augmenté de 50 millions d’euros, passant de 134,7 à 184,4 millions d’euros, alors que les associations chiffrent à 2,6 milliards d’euros le budget minimum que l’État devrait consacrer, chaque année, à la protection des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles en France. Pour l’ensemble de ces raisons,

en 2021, selon l’Insee, 9,1 millions de Français vivaient sous le seuil de pauvreté. Les différentes associations nous alertent sur l’augmentation très importante du nombre de bénéficiaires potentiels de l’aide alimentaire, les femmes et les plus jeunes en première ligne. Avec un budget en augmentation, la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » est donc marquée par un contexte inédit qui nous oblige à intensifier nos efforts auprès des plus fragiles. En effet, au delà des nécessaires solidarité nationale, c’est bien la dignité humaine, dans toutes ses dimensions, qui est en jeu. Nous nous félicitons tout d’abord de la mise en œuvre, cette année, de la déconjugalisation de l’AAH, que le groupe du RDSE avait soutenue et pour laquelle 500 millions d’euros sont prévus en année pleine. Cette réforme concerne 160 000 personnes, dont 80 000 nouveaux bénéficiaires, pour un gain moyen de 300 euros par mois, ce qui n’est pas rien. Nous soutenons pleinement la hausse de 16,26 % des crédits du programme 137 « Égalité entre les femmes et les hommes »,

deux alertes sur des sujets relatifs à nos collectivités locales. La première concerne nos départements, qui se voient confier par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants la mission d’accompagner les jeunes majeurs de moins de 21 ans sortant de l’aide sociale à l’enfance. Il conviendra d’évaluer les effets réels de cette disposition pour les départements, qui indiquent déjà que la dotation prévue, de 50 millions d’euros, ne suffira pas. Ma deuxième alerte concerne le coût de la restauration scolaire supporté par nos communes. L’alimentation des plus jeunes fait partie des priorités que le Gouvernement a mises en avant lors de la présentation du pacte des solidarités pour les années 2024 à 2027. Or l’inflation a touché de plein fouet les tarifs des cantines scolaires et les communes peinent de plus en plus à fournir un prix du repas qui soit acceptable. Le plan prévu il y a un an pour soutenir l’investissement dans les petites communes est il vraiment adapté aux besoins actuels des plus petites collectivités ? Sans doute, madame la ministre, pourrez vous nous éclairer sur son niveau d’exécution budgétaire. Ma dernière remarque concerne les violences faites aux enfants. En France, toutes les trois minutes, un enfant est victime de violences sexuelles. Cette situation est d’autant plus inacceptable et intolérable

Au delà de l’effroi que provoquent ces chiffres, nous savons que nous retrouverons un trop grand nombre de ces enfants marqués par la vie parmi les personnes les plus fragiles et les plus précaires. à lutter contre les violences faites aux mineurs, vient d’être créé au sein de la police judiciaire, ce dont il faut se féliciter. Sa présidente, Gabrielle Hazan, rappelle combien ces violences sont spécifiques et appellent un traitement particulier.

Aussi, mes chers collègues, dans le droit fil des travaux du rapporteur pour avis Laurent Burgoa, je plaide pour qu’une ligne budgétaire dédiée soit consacrée à ce fléau, à l’instar de notre engagement contre les violences faites aux femmes. Le groupe du RDSE votera les crédits de cette mission. La parole

Ces efforts s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été entrepris dans les précédentes lois de finances en matière de politique sociale. Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement demandés sont en hausse de 4,7 % par rapport à la loi de finances initiale Cette mission couvre de nombreux sujets d’importance. En premier lieu, parlons des financements attribués au programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ». Il est essentiel de renforcer les mesures d’aide destinées aux départements, qui font notamment face à une augmentation des dépenses liées à la prise en charge des

Nous nous réjouissons que ce financement soit rétabli ; cela assurera une mise en œuvre pérenne de notre politique d’accompagnement de ces mineurs en situation de précarité. Beaucoup reste à faire, mais par cet amendement, le Gouvernement se tient aux côtés des collectivités territoriales. Nous attendons également

Dans le cadre du pacte des solidarités annoncé le 18 septembre dernier par la Première ministre, les crédits sont mobilisés pour atteindre nos objectifs de sortie de la grande pauvreté. Ces mesures visent particulièrement la prévention de la pauvreté dès l’enfance et l’accompagnement adapté des plus vulnérables vers l’insertion sociale et professionnelle. Ce sont

En deuxième lieu, la mission poursuit les ambitions du plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023 2027, présenté en mars dernier par la Première ministre, en lui allouant des crédits spécifiques. Ceux ci sont destinés à consolider la lutte contre les violences faites aux femmes et à réduire les inégalités sous toutes

Cela représente une augmentation de 20 % des crédits du programme par rapport à la précédente loi de finances. Cette mesure répond avec vigueur aux besoins urgents des victimes de violences conjugales, souvent dans une situation critique pour trouver refuge et rebondir. En troisième lieu, la mission soutient la volonté d’une société plus inclusive, garante de l’émancipation individuelle des personnes handicapées. Je tiens à souligner les efforts faits pour permettre à ces personnes, ainsi qu’aux personnes âgées en perte d’autonomie, de participer pleinement à la société et de choisir librement leur mode de vie. Le développement de l’école inclusive a permis la scolarisation de 430 000 enfants en situation de handicap dans des établissements ordinaires. Divers leviers ont été activés pour soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap, faciliter l’accès aux droits et améliorer la compensation de tous les handicaps. Les crédits alloués au programme « Handicap et dépendance » confirment ces ambitions, en visant notamment à accompagner 21 000 personnes vers l’emploi le dispositif de l’emploi accompagné.

En dernier lieu, la mission s’attache à renforcer les crédits alloués au programme de conduite et de soutien des politiques sanitaires et sociales, avec une augmentation de 22 % des crédits alloués. Parallèlement, ce programme prévoit une hausse de son plafond d’emploi de 41 ETP, ce qui reflète une dynamique positive pour la quatrième année consécutive. Dans ce contexte, le groupe RDPI s’opposera résolument à l’amendement n° II 122 des sénateurs du Rassemblement national visant à supprimer les financements de 630 millions d’euros destinés aux agences régionales de santé (ARS). Cette prise en charge est cruciale pour garantir le bon fonctionnement et la pérennité des emplois au sein de ces structures, qui sont essentielles à notre système de santé. de santé. La mission illustre l’engagement du Gouvernement à garantir l’égalité des chances. Elle démontre l’ampleur des moyens déployés pour continuer les actions de solidarité entreprises ces dernières années. Elle vise enfin à protéger nos concitoyens, dès leur plus jeune âge, de la violence, de la précarité et de l’exclusion. Face à ces enjeux majeurs, le groupe RDPI soutiendra pleinement

la République semblent malheureusement se dissoudre dans une réalité bien plus sombre. Les chiffres sont sans équivoque. D’après la Fondation Abbé Pierre, le nombre de personnes sans domicile fixe a doublé en moins de dix ans, atteignant le seuil critique de 300 000. de victimes de violences conjugales augmente de manière alarmante, avec 244 000 cas recensés en 2022, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. Pauvreté, accès aux soins, inégalités économiques : tous les indicateurs sont au rouge. Les rapports des associations de solidarité résonnent comme des alertes persistantes depuis de nombreux mois, confirmant une augmentation sans précédent de la pauvreté. Selon l’Observatoire des inégalités, 4,8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 1 000 euros par mois. Nous sommes dans une période de régression sociale inquiétante », nous alerte la Défenseure des droits. Les crédits alloués à cette mission devraient combler les besoins des personnes qui restent sur le bord du chemin et qui subissent les insuffisances des politiques de ce gouvernement.

Le budget global de cette mission, qui s’élève à 30,8 milliards d’euros en crédits de paiement, est en augmentation de 4,64 % pour 2024. Il ne répond pas à l’ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » sont ainsi reconduits en 2024. Ce programme couvre principalement la prime d’activité et le RSA recentralisé. Autant dire que cette stagnation du budget n’apportera pas de réponse

grâce à la solidarité à la source pour la prime d’activité et le RSA, l’absence d’augmentation des crédits est incompréhensible, sauf à admettre que votre objectif ne sera pas atteint au détriment, encore une fois, des plus précaires. Je rappelle que le taux de non recours est évalué Ce budget ne suffit pas à compenser l’inflation pour revaloriser le RSA. Les travailleurs et travailleuses précaires sont ceux et celles qui ont recours à l’aide alimentaire,

vous abandonnez la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes au profit d’un pacte des solidarités, avec plusieurs lignes budgétaires en forte régression. Alors que la situation de l’aide sociale à l’enfance est alarmante, des centaines de mesures éducatives ne sont pas mises en œuvre par manque de ressources des associations, de travailleurs sociaux et d’éducateurs. Les associations assurant la protection des majeurs sont très préoccupées par leur incapacité à répondre aux sollicitations. Dans ce contexte, pourquoi diminuer de 6 % la ligne budgétaire pour la protection et l’accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables, alors que les besoins sont criants ? S’agissant du programme 157 « Handicap et dépendance », si des avancées sont à saluer,

Je déplore qu’aucune mesure ne soit prévue pour lutter contre la prostitution, alors que cette réalité sera amplifiée par des événements majeurs tels que les jeux Olympiques et Paralympiques. L’aide financière à l’insertion sociale pour les personnes voulant sortir du système prostitutionnel de 343 euros mensuels est insuffisante pour être efficace. Nous avons déposé un amendement à ce sujet. Nous accueillons favorablement l’aide universelle d’urgence destinée aux femmes pour quitter leur domicile,

à l’ampleur de la situation ! Pour toutes ces raisons, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera contre les crédits alloués à cette mission. La parole

les crédits de cette mission ont progressé de plus de 45 %. Ce n’est donc pas la première année où les politiques de solidarité seront mises à contribution pour répondre à l’urgence sociale. Cependant, le maintien dans le temps long d’une inflation élevée doit nous conduire à une vigilance accrue envers les plus vulnérables, mais également envers ceux qui leur portent assistance. Je pense plus particulièrement aux associations, mais aussi aux départements et aux communes. Ces acteurs sont pris en tenaille entre les demandes d’aide et d’accompagnement qui ne font que s’accroître et l’augmentation de leurs coûts de fonctionnement du fait de l’inflation – plus de 4 % sur les douze derniers mois –, qui touche particulièrement les denrées alimentaires et l’énergie. C’est le cas de l’aide alimentaire, au sujet de laquelle nous partageons la satisfaction du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, Laurent Burgoa, quant au financement supplémentaire qui permettra de soutenir au plus vite la trésorerie des associations concernées. Cependant, nous déplorons que les épiceries sociales et solidaires ne bénéficient que très marginalement de cet abondement. Aussi présenterons nous un amendement de crédits visant à leur consacrer 2 millions d’euros supplémentaires. Au sujet du programme « Handicap et dépendance », nous saluons l’engagement en faveur de l’autonomie des personnes handicapées. Cet engagement se matérialise par l’entrée en vigueur au 1 octobre 2023 de la mesure de déconjugalisation de l’AAH, longtemps soutenue par le Sénat contre l’avis du Gouvernement. Cette avancée pose néanmoins des questions pour l’avenir, notamment lorsque certains des bénéficiaires de l’AAH basculeront vers l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), qui demeure conjugalisée, comme les autres minima sociaux. J’aimerais également souligner les évolutions intervenues concernant les établissements et services d’aide par le travail (Ésat). La mission finance en effet la garantie de rémunération de 120 000 travailleurs en situation de handicap. Les Ésat ont fait l’objet d’un plan de transformation, et plus récemment de mesures dans le cadre du projet de loi pour le plein emploi. Ces évolutions ont permis de renforcer les droits sociaux des travailleurs en Ésat et de les faire converger vers ceux du milieu ordinaire, prise en charge des frais de transport, à la complémentaire santé, aux titres restaurants et aux chèques vacances. Nous nous réjouissons de cet alignement des droits des travailleurs handicapés sur les dispositions du code du travail, qui contribue également à les déstigmatiser. Cependant, ce rapprochement rend urgente l’évolution du modèle financier des Ésat. Laurent Burgoa a souligné dans ses travaux que la mise en place de la seule complémentaire santé représente pour eux une charge de 36 millions d’euros. Or 27 % d’euros. Or 27 % d’entre eux sont déjà déficitaires. Si rien n’est fait pour leur assurer un financement soutenable et pérenne, ces établissements seront obligés de sélectionner les travailleurs handicapés selon leur niveau de productivité, ce qui conduirait mécaniquement à exclure de cet accompagnement des personnes pour lesquelles ce lien avec le monde du travail est pourtant essentiel. Nous appelons donc vivement l’attention du Gouvernement sur ce point et serons vigilants quant aux développements qu’il connaîtra. En somme, nous partageons la conviction d’un besoin de soutien des plus vulnérables face à l’inflation. son poids dans les finances publiques doit nous conduire à suivre avec attention les chantiers qui s’ouvrent en la matière, notamment le déploiement effectif des politiques publiques dans l’ensemble des territoires, y compris dans la ruralité.

les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » recueillent notre assentiment, avec une augmentation – notable, quoique insuffisante – de 4,6 % par rapport à 2023. Nous saluons cette trajectoire, fruit, principalement, de la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés, que nous appelions de nos vœux depuis de nombreuses années. Quand on connaît le retard à rattraper en matière d’égalité des chances et d’inclusion de nos compatriotes en situation de handicap, cette évolution apparaît particulièrement bienvenue. Elle est la réparation d’une injustice qui a trop longtemps eu cours. Cette croissance soutenue des crédits de la mission répond – de manière trop timide, encore une fois – aux profondes difficultés dans lesquelles sont plongés nos compatriotes. À ce titre, les fonds alloués à l’aide alimentaire

Vous avez pourtant refusé la semaine dernière la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, alors que cette mesure, déjà appliquée au Portugal, y a démontré son efficacité. Vous persistez ainsi dans cette politique d’aides ponctuelles, loin de vous approcher d’un changement réel de modèle économique et social et de l’instauration de nouveaux cercles vertueux.

mesure serait pérenne pour nos finances et permettrait d’augmenter directement la rémunération des travailleurs français. Ces crédits représentent ainsi l’écueil principal du Gouvernement : face à la baisse du niveau de vie des Français, il accumule les mesures provisoires et transitoires, cherchant dans des dispositifs conjoncturels des pis aller à la baisse structurelle et constante des revenus, du pouvoir d’achat et de la qualité de vie de nos compatriotes. Néanmoins, dans la démarche de pragmatisme et de poursuite du bien commun qui nous anime, nous saluons l’augmentation des crédits consacrés à l’égalité entre les femmes et les hommes, reposant particulièrement sur une initiative sénatoriale : l’aide exceptionnelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales.

Ainsi, si nous demeurons critiques sur ce budget, sa faiblesse générale et ses péchés originels, nous nous abstiendrons pour ne pas pénaliser les aspects positifs que nous lui reconnaissons. La parole

Monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues, pour 2024, les crédits demandés pour la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » s’élèvent à 30,85 milliards d’euros, soit 4,64 % de plus par rapport à 2023. Cette hausse est essentiellement due à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prime d’activité, qui représentent à elles seules 78,5 % des crédits de la mission. Parmi les nouveaux apports de crédits, 13 millions d’euros sont attribués à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales. Issue d’une proposition de loi du Sénat, cette mesure permettra aux victimes de bénéficier d’une petite aide financière. Je souhaite néanmoins souligner que les associations qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales manquent cruellement de moyens et que la permanence qu’elles assurent est menacée, notamment en milieu rural. La déconjugalisation de l’AAH, entrée en vigueur le 1 octobre dernier, permettra à 40 000 personnes de bénéficier d’une augmentation de leur allocation et étendra le dispositif à 80 000 autres personnes. Le coût de cette mesure représentera 500 millions d’euros Autre évolution très significative, les crédits consacrés à l’aide alimentaire augmenteront de 20,6 %, pour un total de 142 millions d’euros. Cette augmentation, qui a le mérite d’être importante, risque toutefois d’être insuffisante. Les banques alimentaires font en effet part de leurs inquiétudes depuis plusieurs mois sur les difficultés auxquelles elles font face en matière d’approvisionnement de denrées, notamment de la part de la grande distribution. À cela s’ajoute l’explosion du nombre de demandeurs. Dans mon territoire par exemple, le Maine et Loire, les Restos du Cœur distribuaient au début des années 2000 environ 800 000 repas par an. Aujourd’hui, c’est un million de plus ! Et cette évolution s’illustre bien plus largement sur tout le territoire national. La véritable solution est de permettre à chacun de nourrir sa famille, en vivant dignement de son travail. C’est la raison pour laquelle notre groupe avait unanimement soutenu le projet de loi pour le plein emploi. Il permettra un meilleur accompagnement des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du RSA, à condition de donner à France Travail et aux départements les moyens de la mise en place de cette réforme. Le programme « Handicap et dépendance » prévoit 1,61 milliard d’euros afin de garantir la rémunération des travailleurs en Ésat. Nous soutenons cette mesure.

Enfin, comme d’autres sénateurs, je me suis étonnée de la baisse des crédits alloués aux départements et consacrés aux MNA. Cette baisse était d’autant plus étonnante qu’elle est en rapport avec les effets attendus d’un projet de loi sur l’immigration qui n’est pas encore adopté adopté et alors que les départements sont déjà pris à la gorge d’un point de vue financier. L’amendement du Gouvernement relevant le niveau de ces crédits est donc bienvenu.

Je tiens à remercier notre collègue rapporteur pour avis Laurent Burgoa pour son travail sur les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Cette mission est destinée à lutter contre la pauvreté, à réduire les inégalités et à protéger les personnes vulnérables. en hausse de 4,64 % par rapport à 2023, s’explique par la revalorisation des prestations sociales et de l’aide alimentaire pour faire face au défi de l’inflation. Nous y sommes favorables, puisque la crise inflationniste nécessite des mesures gouvernementales de soutien pour les ménages les plus précaires. La mission comprend quatre programmes. Le programme « Égalité entre les femmes et les hommes » ouvre les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, Nous nous félicitons de l’entrée en vigueur de ce dispositif. J’ai eu le plaisir d’être rapporteure de ce texte et je suis heureuse de voir sa concrétisation : cette loi offre aux femmes victimes de violences conjugales l’espoir d’un nouveau départ. L’amendement II 687 rectifié de Dominique Vérien et des membres du groupe Union Centriste vise à améliorer les modalités de remboursement de cette aide par les bénéficiaires.

la prime d’activité, inscrite dans le programme « Inclusion sociale et protection des personnes », et l’allocation aux adultes handicapées dans le programme « Handicap et dépendance ». Compte tenu de l’augmentation sensible du nombre des bénéficiaires, la hausse des crédits permettrait de répondre à l’urgence sociale. Nous saluons l’entrée en vigueur de la déconjugalisation de l’AAH, tant attendue par les personnes en situation de handicap et fortement soutenue par le Sénat. Cette avancée permettra à 40 000 bénéficiaires en couple de voir leur allocation augmenter et à 80 000 nouvelles personnes de bénéficier de cette allocation. Nous resterons vigilants sur un point particulier : en effet, la déconjugalisation de l’AAH risque d’entraîner des décrochements de revenus dans les parcours de vie de certains bénéficiaires. C’est le cas notamment de ceux qui bénéficient de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui, elle, n’est pas déconjugalisée. Ce sujet est à approfondir pour l’avenir. Nous sommes aussi favorables aux deux articles additionnels rattachés à la mission, retenus par le Gouvernement. L’un permet aux bénéficiaires de l’AAH de continuer à percevoir leur allocation, s’ils décident de poursuivre leur activité après avoir atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite. L’autre prévoit le maintien pour les bénéficiaires de l’AAH des prestations liées – majoration pour la vie autonome et complément de ressources –, lorsqu’ils perdent le bénéfice de l’AAH du fait de la revalorisation de leur pension. La mission contient également des mesures de transfert, notamment concernant les moyens dédiés aux prestations d’aide sociale à destination des personnes sans domicile fixe âgées ou en situation de handicap. de handicap. Les différentes associations de solidarité, mais aussi les départements, témoignent d’une augmentation des demandes d’aides et d’accompagnement. Cela mettra en péril l’autonomie financière des départements. En ce qui concerne la compensation aux départements des frais relatifs à la mise à l’abri et à l’évaluation des mineurs non accompagnés, les crédits prévus sont en retrait de 22,1 millions d’euros. Cette diminution est justifiée par l’impact du projet de loi sur l’immigration sur les flux de MNA. Cette estimation nous semble, à ce jour, pour le moins optimiste et une telle décision risque de mettre de nouveau en difficulté la trésorerie des départements. Par ailleurs, l’obligation des départements d’accompagner les jeunes majeurs de moins de 21 ans sortant de l’aide sociale à l’enfance sera compensée par un abondement de 50 millions d’euros en faveur des collectivités. Ce montant paraît déconnecté de la charge réelle, puisque les départements constatent déjà une augmentation de 15 % de cette dépense. Force est de constater que le manque de moyens alloués à la protection des personnes, majeures comme mineures, risque de poser de réels problèmes aux collectivités territoriales et aux associations concernées. Concernant la prévention et la lutte contre la pauvreté, le pacte des solidarités succède à la stratégie nationale 2018 2022. Doté de 260 millions d’euros sur le périmètre de la mission, il comporte quatre axes pour réduire les inégalités dès l’enfance, amplifier l’accès à l’emploi pour tous, lutter contre l’exclusion grâce à l’accès aux droits et construire une transition écologique solidaire. Nous saluons ces engagements, notamment parce que « le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion », pour reprendre les mots de Victor Hugo. Nous nous interrogeons néanmoins sur la portée réelle de ce plan. En outre, nous regrettons le manque de lisibilité qui résulte de l’éclatement des financements de ce pacte entre plusieurs missions. Cependant, nous sommes satisfaits de la poursuite de la pratique de contractualisation avec les collectivités territoriales pour lutter contre les pauvretés. Les crédits consacrés à l’aide alimentaire connaissent une augmentation, mais cela ne répond qu’imparfaitement aux besoins liés à une inflation élevée sur les denrées alimentaires.

Enfin, grâce au programme « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », les agences régionales de santé voient leur subvention pour compensation d’obligations de service public augmenter afin de financer de nouveaux recrutements dans les secteurs de l’autonomie et du handicap. Nous saluons ces créations de postes, mais nous nous interrogeons sur leur pérennité, compte tenu du déficit d’attractivité dont souffre le secteur social. Vous l’aurez compris, le groupe Union Centriste soutiendra les crédits de cette mission, sous réserve de l’adoption de l’amendement déposé par la commission des affaires

la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » du projet de loi de finances pour 2024 concerne les politiques en faveur des personnes les plus fragiles, particulièrement les politiques de l’emploi, du handicap, de la protection de l’enfance et de lutte contre les violences faites aux femmes.

sont liées au revenu de solidarité active ou à la prise en charge des mineurs non accompagnés. Comme vous le savez, mesdames les ministres, plusieurs départements ont annoncé suspendre ou limiter les prises en charge, faute de moyens et de personnel encadrant. En tant que conseillère d’Alsace, je connais cette saturation du dispositif due à l’augmentation constante des flux. Actuellement, la Collectivité européenne d’Alsace

compétence régalienne de l’État. Dans ce domaine, il faut agir vite, mesdames les ministres, car la situation n’est pas humainement tenable. De façon plus générale, l’insuffisance des crédits consacrés à la protection et à l’accompagnement des enfants risque, selon le constat de notre rapporteur pour avis Laurent Burgoa, de conduire à des situations de maltraitance institutionnelle. C’est inacceptable au regard de la situation alarmante décrite très récemment par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants son rapport rendu public le 17 novembre. Alors qu’on recense 160 000 victimes par an, 70 % des plaintes sont classées sans suite. Cette commission a effectué un travail considérable pour alimenter les décisions gouvernementales et leur mise en œuvre, du repérage des maltraitances au traitement judiciaire, en passant par la prise en charge des soins et de la prévention. Ne pas suivre ses recommandations, faute de moyens, serait réellement irresponsable. Nous serons donc attentifs

L’émancipation économique des femmes devrait être une priorité politique et collective. Or nous constatons l’inverse dans les faits : pénalisées sur le marché du travail par leur statut d’aidant à tous les âges de la vie, par les congés maternité et les emplois précaires, qu’elles occupent davantage que les hommes, les femmes subissent une violence économique qui ne fait que s’aggraver. Ces inégalités se cumulent et ont des répercussions sur le montant de leur retraite, qui, je le rappelle, est inférieur de 40 % en moyenne à celui des hommes. Là encore, mesdames les ministres, il faudra impérativement corriger cet état de fait et repenser la dépendance économique des femmes,

ainsi que « le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Pourtant, en France, selon l’Unicef, un enfant sur cinq, soit près de 3 millions d’enfants, vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2018. L’annexe budgétaire de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances

Selon le plan national nutrition santé, le petit déjeuner est un repas à part entière et doit représenter entre 20 % et 25 % des apports énergétiques de l’ensemble d’une journée. Or la prise du petit déjeuner n’est pas systématique chez les enfants.

du programme 304

à ceux de l’ancienne action n° 19, qui concernait la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, dotée de 257 millions d’euros. Le pacte des solidarités du Gouvernement n’est doté que de 190 millions d’euros. prévoit donc une baisse des crédits destinés à la lutte contre la pauvreté de 60 millions d’euros, dans un contexte où la pauvreté touche 9,2 millions de personnes, soit près de 15 % de la population. Alors que l’ensemble des associations de solidarité alertent depuis plusieurs mois sur les difficultés qu’elles rencontrent du fait du nombre grandissant de bénéficiaires, c’est un très mauvais signal qui leur est adressé.

Le Gouvernement a annoncé en septembre 2023 son pacte des solidarités, qui vise à « contenir la pauvreté », pour reprendre les termes de la Première ministre. Selon le collectif Alerte, qui rassemble associations, il s’agit plus d’un plan de gestion de la pauvreté que d’un plan de lutte contre la pauvreté. Ces éléments démontrent la volonté gouvernementale de ne pas agir efficacement

précis. Elle souhaite en effet encourager le plus possible le recours à la contractualisation avec les collectivités territoriales pour la mise en œuvre du pacte des solidarités. Or le présent amendement semble donner un blanc seing au Gouvernement et allouer 10 millions d’euros supplémentaires aux actions pilotées par l’État, alors qu’un fléchage vers les collectivités et les besoins sur le terrain devrait être recherché. À titre personnel, j’émettrai toutefois un avis favorable

Le droit à la dignité et la protection de l’intérêt supérieur de ces enfants ne peuvent être garantis dans la rue. La baisse des températures fait peser un risque supplémentaire sur leur santé. Aucun enfant ne peut être abandonné dans nos rues. Il convient donc d’abonder significativement les crédits de la politique relative à l’hébergement d’urgence des enfants et de leurs parents, afin de ne pas séparer les familles, en conformité avec leur droit au respect de la vie privée et familiale. Cet amendement vise à prévoir 7 millions d’euros afin de financer un mois d’hébergement d’urgence pour 2 800 enfants et un parent.

Mais nous sommes démunis face à cet amendement, car il concerne une politique, celle du logement et de l’hébergement d’urgence, qui ne relève pas de la mission « Solidarité,

Une forte mobilisation des élus locaux a permis de convaincre le Gouvernement de renoncer à la fermeture de 14 000 places d’ici l’année prochaine et de stabiliser le parc d’hébergement, cela n’est pas suffisant. Selon une note d’analyse de la Fédération des acteurs de la solidarité, les niveaux de financement des centres d’hébergement d’urgence convergent autour de 27 euros par jour et par Étant donné que la France compte 300 000 personnes sans domicile fixe, l’adoption de cet amendement nécessiterait l’abondement de sommes considérables dans un programme consacré au sans abrisme.

par la création d’un fonds spécifique de prise en charge des psychotraumatismes causés aux enfants. Chaque année, en France, au moins 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles.

d’une Uaped par juridiction. La participation de l’État pour chaque unité est de 60 000 euros. Les 7,4 millions d’euros fléchés dans le cadre du PLF pour 2024 sont donc insuffisants

vise à entériner l’annonce récente faite par le Gouvernement sur la poursuite du travail de la Ciivise avec « des modalités et une feuille de route renouvelées et centrées sur de nouvelles missions ».

je profite de cet amendement pour appeler de mes vœux le maintien dans ses fonctions du juge Durand, ce qui est le souhait manifeste de l’ensemble des associations. je vous propose d’abonder de 2 millions d’euros l’action n° 17 « Protection et accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables », afin de rendre effectif le maintien de la Ciivise.

Nous considérons, comme les nombreux signataires de la tribune parue en septembre dans le journal, que la Ciivise est éminemment utile et que son mandat devrait être prolongé. Le Gouvernement peut il garantir à la représentation nationale la pérennité de l’existence de cette commission ? Quel est l’avis du Gouvernement ? Merci, mesdames,

Cette démarche doit être valorisée et ne peut pas être absorbée, noyée, effacée dans des questions budgétaires. Ce que ces militants

Cet amendement concerne un sujet d’une urgence sociale et humaine profonde : le soutien aux familles des enfants devenus orphelins à la suite d’un féminicide. Depuis 2011, plus de 1 200 enfants sont devenus orphelins après la perte tragique de leur mère, victime d’homicide conjugal – ce sont majoritairement des féminicides. Ces familles déjà frappées par un traumatisme inimaginable sont doublement affectées, lorsqu’elles doivent assumer, en plus, la charge financière de ces enfants endeuillés. L’amendement que je propose vise à créer un programme spécifique de soutien à ces familles au sein de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », avec une dotation initiale de 2 millions d’euros. Cette initiative, qui est un geste de solidarité et de responsabilité envers les plus vulnérables de notre société, serait financée par un redéploiement des crédits de l’action n° 11 du programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

La situation des familles devant prendre en charge ces orphelins est également difficile – personne ne le nie. Toutefois, la commission peine à déterminer comment le présent amendement peut apporter une réponse satisfaisante à ces difficultés. Rapporté aux 1 200 enfants concernés chaque année, le montant proposé de 2 millions d’euros représenterait 1 666 euros par enfant. Si ce soutien vise à dédommager les familles et l’enfant,

Parmi les 118 victimes de féminicide en 2022, 37 avaient déjà subi précédemment des violences par leurs conjoints ou ex conjoints, 24 les avaient signalées aux forces de l’ordre, 16 avaient déposé des plaintes. Elles ont pourtant rejoint le cortège des disparues sous les coups de ceux qui préféraient les voir mortes plutôt que libres. Réduites au silence, elles avaient pourtant parlé pour dénoncer les violences dont elles étaient les victimes. Les enfants, eux aussi, sont des victimes directes. À ce titre, la commission de violences intrafamiliales doit être prise en compte pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

La Fondation des femmes a évalué à 2,6 milliards d’euros le budget nécessaire pour éradiquer les violences patriarcales. Nous devons, à la mémoire des trop nombreuses victimes, l’engagement ferme et entier de toute la société dans un seul but : éradiquer les violences faites aux femmes.

Au sein du décompte glaçant du collectif « Féminicides par compagnons ou ex », les enfants covictimes de meurtres conjugaux sont régulièrement cités parmi les disparus. Les écoutants du 119 témoignent de conditions de travail dégradées en raison d’un flux d’appels trop nombreux, que les effectifs actuels ne permettent pas d’absorber. Pour certains, le 119 sauve des vies ; pour d’autres, la ligne ouvre une porte vers la fin des violences et des maltraitances.

permettraient aux pouvoirs publics de disposer plus rapidement des données nécessaires à l’accomplissement de leur mission de protection de l’enfance en danger. En effet, à la suite de l’audition de la France dans le cadre de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant,

le pilotage d’une politique publique adéquate susceptible de résorber les retards significatifs d’exécution. On constate que, dans certains départements, plusieurs mois s’écoulent entre le prononcé

beaucoup plus rapidement entre la décision et l’exécution.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

et violentes. En créant un référent national du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) affilié à France Enfance protégée, nous renforcerions les procédures de vérification des antécédents des professionnels qui sont en contact avec les mineurs.

contribuerions ainsi à garantir un environnement sûr pour les enfants. Cet amendement prévoit donc un abondement de 120 000 euros du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes ». Un prélèvement équivalent sur le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales » garantirait une redistribution

Cet amendement vise à accorder une allocation supplémentaire de 60 millions d’euros aux associations d’aide alimentaire. Ces associations ont tiré la sonnette d’alarme et mis en évidence leur fragilité persistante.

une mesure d’urgence qui ne résout en rien le problème structurel de l’insécurité alimentaire touchant des millions de Français. Les 60 millions d’euros supplémentaires que nous proposons permettraient à ces associations de répondre de manière plus adéquate aux besoins grandissants, à l’inflation, mais aussi à l’augmentation du nombre de bénéficiaires. Quel

Néanmoins, elle appelle de ses vœux une augmentation équivalente de son volet national. En effet, ce volet concerne les approvisionnements des associations d’aide alimentaire, tandis que le volet local finance avant tout des projets et nouvelles démarches sélectionnés au travers d’un appel à projets.

ce programme a été doté en 2023 de 60 millions d’euros, puis de 70 millions d’euros pour 2024. Une augmentation de 10 millions d’euros a donc déjà eu lieu. En outre, si l’objectif de cet amendement est de répondre à l’urgence sociale, il convient de relever que le programme « Mieux manger pour tous » n’est pas l’instrument idoine. En effet, les acteurs associatifs ont relevé l’inadéquation de ce programme avec les besoins conjoncturels très forts du secteur. Certes, il s’agit d’une initiative louable pour transformer structurellement et sur le long terme l’offre d’aide alimentaire, mais elle n’est pas adaptée pour répondre à l’urgence, ne serait ce que parce que les produits bio et locaux sont chers, en période de

d’actions d’information et de soutien aux tuteurs familiaux. Lors des travaux de la commission, les représentants de ce secteur ont souligné la forte dynamique du nombre des mesures de protection prononcées par les juges des tutelles, notamment du fait du vieillissement de la population. En effet, un million de personnes vulnérables bénéficient d’une mesure de tutelle ou de curatelle, en raison de l’altération de leurs facultés personnelles, qui rend indispensable leur assistance ou leur représentation dans les actes de la vie civile.

Lors de nos auditions, les associations du secteur du handicap ont indiqué qu’aucun financement ne semblait prévu pour poursuivre et renforcer la dynamique du Fatésat. Pourtant, une enveloppe de 15 millions d’euros a été envisagée lors du premier comité de suivi du plan de transformation des Ésat.

entre les aidants et leurs proches en situation de handicap, de maladie chronique ou de perte d’autonomie liée à l’âge. Ces solutions prennent tout particulièrement la forme de résidence de répit partagé relevant du code de l’action sociale et des familles. Une résidence de répit partagé propose un accueil temporaire à vocation médico sociale de la personne aidée en présence d’un ou plusieurs aidants familiaux, tout en leur offrant conjointement des prestations de tourisme

Il existe en effet plus de 11 millions d’aidants familiaux en France, soit un Français sur cinq ! Sept aidants sur dix refusent l’idée d’un placement définitif de leur proche aidé et aspirent à ce qu’un droit au répit partagé soit effectif. Plus d’une dizaine de territoires, avec l’appui notamment des conseils départementaux, qui sont toujours en lien avec les associations représentatives des personnes et des aidants, sont porteurs de ces projets novateurs de résidence de répit partagé.

à financer les acteurs proposant des séjours de vacances pour favoriser le répit des aidants. D’une part, le financement d’acteurs touristiques n’est pas habituel pour les ARS, qui évoquent des risques vis à vis du droit de la concurrence.

pour accueillir des personnes dépendantes, handicapées ou âgées avec leur accompagnant. Certes, évidemment, la zone choisie est agréable, donc un peu touristique, mais il n’y a aucun rapport avec une résidence touristique. Madame la ministre, l’année dernière,

Pour mémoire, plus de 800 000 femmes sont chaque année écoutées, accompagnées, hébergées et soutenues au sein des centres d’accueil de jour spécialisés, des lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation (LEAO) ainsi que des permanences juridiques et sociales partout en France. Quel

Il convient également de noter que les sommes demandées dans cet amendement équivalent à près du quart des crédits du programme, qui ont déjà connu une progression importante ces dernières années, et qui augmentent encore de 22 % dans le budget 2024. Nous demandons donc le retrait de cet amendement. Quel est l’avis du Gouvernement ? Je suis très

des signalements, le budget prévu par le Gouvernement ne permet pas de répondre, de manière efficiente, à chaque dénonciation, à chaque alarme, à chacun des signaux faibles que les pouvoirs publics et les associations doivent pourtant saisir

voient souvent obligées de dégrader la qualité de leur offre. En pratique, cela signifie, par exemple, que des victimes n’auront pas d’autre solution que de retourner chez leur conjoint violent

certaines associations, malgré leur diligence et leur bonne volonté, peinent à obtenir des services de l’État le versement en temps et en heure des aides qui pourraient leur permettre de se développer. Bien souvent, celles ci ne perçoivent qu’en fin d’année fin d’année les subventions pour lesquelles elles se sont parfois portées candidates en début d’année. Il nous semble qu’il faudrait commencer par régler la question du conventionnement et des avances en cours d’année pour que les réponses soient, en termes de calendrier, cohérentes avec les décisions. demande le retrait

pour une personne seule, n’est toutefois pas suffisant, d’autant qu’elle est limitée dans le temps. Aussi, cet amendement tend à augmenter le montant de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle, afin d’accompagner au mieux les personnes qui le souhaitent dans une sortie durable du parcours prostitutionnel. L’amendement

Ce faisant, un éclairage cru a été apporté à la réalité des violences sexuelles et des tortures infligées aux femmes dans l’industrie pornographique. Plusieurs victimes sont engagées dans des démarches d’ordre judiciaire ou non, que ce soit pour faire reconnaître les violences qu’elles ont subies ou pour faire valoir leurs droits à l’oubli

interdit l’achat d’actes sexuels. Cette interdiction envoie un message clair aux clients et aux proxénètes : le corps des femmes n’est pas à vendre. Il s’agit d’un pilier essentiel de la politique abolitionniste de la France. L’organisation d’événements sportifs internationaux d’envergure comme les jeux Olympiques a des conséquences sur le trafic des êtres humains, car elle incite les réseaux de proxénétisme à déployer leurs efforts

pour le déploiement d’une campagne de communication à la hauteur des enjeux. qui accompagnera immanquablement les jeux Olympiques risque fort de diluer le message porté par une telle campagne. Il semble qu’il s’agisse de nouveau d’un amendement d’appel dont nous demandons le retrait. Cela étant, nous entendrons avec beaucoup d’intérêt le Gouvernement, parce qu’évidemment le problème soulevé

Si la commission s’interroge sur l’opportunité de décider d’une subvention à accorder à une association précise, ce qui n’est pas dans nos habitudes, elle s’en remet toutefois à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

que nous avons décidé d’augmenter significativement les moyens du 3919 2,9 millions d’euros , justement pour accompagner les écoutants, mais aussi pour déployer

Miquelon. Quel est l’avis de la commission ? au vu de l’expérience passée, il ne semble pas nécessaire d’y allouer davantage de crédits.

Merci,